J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

En outre, de nouveaux enjeux se font jour pour les territoires d’outre mer, dont les crédits de la mission devront tenir compte à l’avenir. En effet, la crise sanitaire a souligné la très grande dépendance des territoires ultramarins aux importations alimentaires,

À cet égard, les annonces faites à l’issue du comité interministériel des outre mer (Ciom) de juillet 2023 représentent une avancée notable, sans répondre néanmoins à toutes les attentes. Reste surtout à les concrétiser par des moyens budgétaires et par un réel suivi, régulier et exhaustif.

Force est cependant de constater que, si des annonces ont été faites en ce sens lors du Ciom, aucune mesure d’ensemble sur le pouvoir d’achat n’a été actée.

est du programme 123, qui recense les crédits des politiques publiques en faveur de l’amélioration des conditions de vie dans les outre mer, cette hausse porte sur trois domaines fondamentaux pour nos territoires. Tout

En revanche, les crédits alloués à l’appui à l’accès aux financements bancaires et au soutien en ingénierie diminuent, alors même que le besoin de financement des acteurs économiques locaux pourrait augmenter en 2024, dans un contexte de crise économique.

d’autre part, les crédits alloués au fonds outre mer aux fins de développer le soutien à l’ingénierie des communes et intercommunalités de Polynésie. Ce second point comptait du reste au nombre des préconisations de notre rapport sur les Corom. outre mer », qui rassemble les crédits des politiques publiques en faveur de la compétitivité des entreprises, de l’amélioration de l’employabilité des jeunes et de la qualification des actifs ultramarins, il enregistre également une hausse substantielle. Cette hausse résulte essentiellement de celle des crédits consacrés aux exonérations de charges sociales, dans un contexte où la masse salariale en outre mer augmente régulièrement depuis 2022 et la fin de la crise sanitaire.

je salue bien entendu, comme mon collègue Georges Patient, la hausse des crédits de la mission « Outre mer ». Il convient également de rappeler que ces crédits ont, de surcroît, été augmentés par plusieurs modifications apportées par l’Assemblée nationale. Je pense notamment à la hausse du fonds exceptionnel d’investissement

et à l’effort général de rattrapage de l’écart de niveau socioéconomique entre l’outre mer et la métropole. Les dépenses fiscales associées aux deux programmes de la mission devraient s’établir, en 2024, à plus de 5 milliards d’euros, soit deux fois plus que les crédits budgétaires portés par la mission elle même. pour 2023, plusieurs modifications bienvenues étaient intervenues pour prolonger, jusqu’en 2029, des dépenses fiscales dont le fait générateur allait s’éteindre. Je me souviens également d’un amendement adopté par le Sénat qui étendait le bénéfice de ces dispositions aux collectivités du Pacifique. Nous estimons que ces dépenses fiscales sont un outil indispensable pour l’économie ultramarine, tout en reconnaissant qu’il est nécessaire de mieux les évaluer et, au besoin, de les modifier. Dans ce contexte, les démarches entreprises ces dernières années vont dans le bon sens et doivent être poursuivies.

L’acceptabilité et la pertinence de ces réformes dépendront du dialogue qui sera mis en place. Les débats intervenus dans notre assemblée en première partie, notamment sur l’article 7 , témoignent de la nécessité d’adapter la méthode.

d’engagement et de 648 millions d’euros en crédits de paiement. Ces crédits pluriministériels permettent, notamment, le financement de plusieurs plans thématiques importants pour nos territoires d’outre mer : le plan d’actions pour les services d’eau potable et d’assainissement, le plan Séisme Antilles, le plan Sargasses, le plan Logement outre mer et le plan Chlordécone. Nous saluons donc leur augmentation. Enfin, les territoires d’outre mer bénéficient des crédits du plan de relance et du fonds vert.

Cette sous consommation, en deçà des attentes et en deçà des besoins, s’explique pour partie par la faiblesse de l’ingénierie en outre mer et par d’autres contraintes locales, comme la difficulté à trouver du foncier disponible.

S’il en était besoin, la mise en œuvre du plan de relance, comme celle d’autres dispositifs auparavant, met en exergue l’absolue nécessité de tenir compte des spécificités territoriales et de développer des approches différenciées entre la métropole et les territoires d’outre mer, mais également entre les territoires d’outre mer eux mêmes. mes chers collègues, il s’agit tout simplement de tenir compte des lois organiques portant statut de nos territoires respectifs votées par le Parlement national. Le fonds vert, pour sa part, a été fortement sollicité en outre mer. Ainsi, 403 dossiers ont été déposés

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a choisi de rendre un avis favorable sur les crédits de la mission « Outre mer » pour 2024. 2024. Les crédits dédiés aux territoires ultramarins étant répartis au sein de trente deux missions budgétaires, c’est peu dire qu’il n’est pas aisé d’apprécier dans sa globalité l’effort consenti par l’État en faveur du rattrapage de nos territoires ultramarins. Pour ce qui est des crédits du très restreint périmètre de la mission « Outre mer », nous notons avec satisfaction que nombre des recommandations de notre assemblée, portant notamment sur le logement ou sur la continuité territoriale, ont été suivies dans le cadre de ce budget, ainsi que dans celui des annonces issues du comité interministériel des outre mer. Naturellement, beaucoup reste à faire ; mais, lorsque le Gouvernement reprend à son compte des propositions qui lui sont faites, il convient de le noter. ce qui concerne la question du logement social, sur laquelle je souhaite insister, les résultats en matière de construction, de réhabilitation et de lutte contre l’habitat indigne demeurent très en deçà des ambitions affichées, année après année, par le Gouvernement. Avec 2 729 logements livrés en 2022, nous avons atteint un point bas historique de la construction, alors que 80 % des ménages ultramarins sont éligibles au logement social. Le rythme des réhabilitations, environ 2 000 par an, n’est pas non plus satisfaisant, au regard des besoins observés et du vieillissement de certaines populations que l’on entend maintenir à domicile. Enfin, que dire de la lutte contre l’habitat indigne ? ? Près de 150 000 logements indignes sont recensés par la Fondation Abbé Pierre et près de trois Ultramarins sur dix seraient en situation de mal logement ou confrontés à l’absence de logement personnel, ce qui témoigne, monsieur le ministre, de l’insuffisance de votre politique.

qui intervient dans un contexte encore incertain pour les territoires ultramarins, marqué par une inflation persistante, une aggravation des inégalités et une multiplication des tensions sociales. Ces crédits supplémentaires permettront, tout d’abord, de financer la construction de logements et la lutte contre l’habitat indigne, qui constituent un enjeu majeur. Vous le savez, les logements insalubres représentent en moyenne 18 % des logements en outre mer. Ces crédits permettront, ensuite, le renforcement de la continuité territoriale, notamment grâce à l’élargissement des publics éligibles à l’aide à la continuité territoriale. Les ouvertures de crédits ont également vocation à renforcer l’insertion professionnelle, par exemple la poursuite du déploiement du plan SMA 2025+, qui vise à améliorer le service militaire adapté, dont l’efficacité n’est plus à prouver. au soutien aux collectivités territoriales, il sera renforcé : en témoignent la pérennisation des contrats de redressement en outre mer et le financement de nouveaux contrats de convergence et de transformation. Si cette hausse des crédits est bienvenue, je souhaiterais toutefois insister sur deux points. Tout d’abord, il est indispensable de poursuivre cet effort budgétaire dans la durée, notamment dans le domaine du logement, afin de fournir un habitat décent à chaque citoyen ultramarin.

Toutefois, la gestion de la mission reste marquée par une sous consommation des crédits, qui concerne notamment la ligne budgétaire unique. Compte tenu de l’ampleur des enjeux relatifs à l’habitat insalubre en outre mer,

concernant la compensation des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises ultramarines. Enfin, le volume de restes à payer, qui est très élevé, représente un risque avéré pour la soutenabilité de la mission budgétaire. La commission des lois appelle donc le Gouvernement à poursuivre l’amélioration du pilotage budgétaire de la mission. En dépit de ces quelques faiblesses, et compte tenu des éléments positifs

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour 2024, les moyens financiers déployés en faveur de la mission « Outre mer s’élèvent à 2,9 milliards d’euros en autorisations d’engagement et à 2,6 milliards d’euros en crédits de paiement à périmètre constant, soit des hausses respectives de 6,8 % et de 4,5 % par rapport à 2023. et indépendants salue cette augmentation des moyens au service de nos concitoyens. La mission « Outre mer » répond à quatre grandes orientations budgétaires de la politique du Gouvernement.

qui concerne le logement, l’augmentation de la ligne budgétaire unique permettra de financer les grands défis de nos territoires, à savoir la construction de logements locatifs sociaux, la réhabilitation et l’adaptation au vieillissement du parc locatif parc locatif social, sans oublier la lutte contre l’habitat indigne. Concernant ensuite l’accès à l’eau, nous saluons la pérennisation du soutien apporté au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, à hauteur de 20 millions d’euros.

La deuxième orientation du budget vise à accompagner la mobilité des Ultramarins. Rappelons le contexte : les Ultramarins pâtissent d’une hausse substantielle et continue du prix des billets d’avion depuis deux ans.

Une augmentation de 57,5 % du tarif des billets d’avion a même été enregistrée au départ de la Martinique en mars 2023, selon la

Ces moyens supplémentaires permettront de relever le seuil d’éligibilité aux aides de Ladom – merci pour les étudiants et merci pour tous ceux qui partent en formation ! Il nous reviendra également d’examiner l’évolution des dispositifs d’accompagnement des professionnels à la mobilité. Or je sais pouvoir compter sur l’engagement et la mesure de la Haute Assemblée pour aboutir à la meilleure solution pour nos outre mer.

ce dispositif n’est pas accessible aux communes dans le Pacifique. C’est pourquoi je salue l’amendement déposé par Teva Rohfritsch pour soutenir les communes polynésiennes. En outre, dans la continuité de ses efforts budgétaires, l’État poursuit son accompagnement à la collectivité territoriale de Guyane.

faut un contrôle ! Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera les crédits de cette mission. La parole

qu’il en soit, ce rapport et cet amendement sont malheureusement symptomatiques de la façon dont Bercy considère nos territoires, nos élus et nos acteurs économiques. La réforme des aides économiques engagée dans le PLF pour 2019 était pourtant un cas d’école.

à chacun d’entre eux. Le « réflexe outre mer », c’est considérer l’outre mer dans sa singularité ; c’est aussi admettre que cette singularité s’apprécie territoire par territoire

C’est un levier évident ; et pourtant nous ne pouvons en bénéficier. Les exemples de ce type ne manquent pas. Trop de lois et de décrets sont source de blocages qui entravent le travail de nos collectivités.

on entre en dépendance aux alentours de 65 ans, contre 85 ans en métropole, et la plupart des personnes dépendantes souhaitent rester à domicile. La Réunion s’est fortement impliquée

Au cours de ce débat, je défendrai un amendement visant à allouer 250 000 euros à la réalisation d’enquêtes locales et au soutien aux associations luttant contre les violences faites aux enfants dans les outre mer. qui est de l’article 55, il importe de garantir la sélection des projets professionnels en fonction des besoins réels des territoires ; monsieur le ministre, pourriez vous nous fournir une ébauche d’éléments méthodologiques à ce sujet ?

Grâce à eux, à nos 2 millions de compatriotes qui y vivent, à la formidable diversité de leurs ressources et de leurs talents, la France dispose du deuxième espace maritime mondial et d’une présence globale à même d’asseoir son rôle de partenaire incontournable dans un monde changeant.

du manque de services ou de l’abandon par l’État des collectivités territoriales, l’outre mer appelle au secours et le Gouvernement reste sourd. Quelle vision l’exécutif nous présente t il avec la mission « Outre mer » ? Aucune.

À La Réunion, la crise du logement est telle que les services de l’État estiment à 40 000 le nombre de logements nouveaux manquants pour nos compatriotes. En Guyane, l’immigration irrégulière et l’orpaillage illégal terrifient les habitants. Profitant de l’inflation, le Gouvernement annonce une augmentation minime du budget de la mission « Outre mer » : dont acte. Mais ces quelques millions d’euros saupoudrés ne permettront en rien d’atténuer le sous développement structurel de nos territoires ultramarins. Ainsi, monsieur le ministre, vous ne revenez pas sur le régime de l’octroi de mer, imposition anachronique qui renchérit de 20 % le coût de la vie. Vos efforts en faveur de l’autonomie alimentaire et énergétique de ces territoires ne sont que de vagues promesses. Face à la décrépitude des services publics les plus élémentaires, votre ministre de tutelle invite les Mahorais à faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire. Vous faites maintenant rimer incompétence avec indécence. tel budget n’assure ni l’ordre, ni le développement, ni le respect de la dignité de nos départements et territoires d’outre mer. Les élus du Rassemblement national voteront donc contre les crédits de cette mission. Nous nous inclinons devant l’infinie patience de nos compatriotes ultramarins devant cette situation indigne cultivée depuis trop longtemps.

À cette fin, le programme « Emploi outre mer » est doté de 1,86 milliard d’euros en autorisations d’engagement et de 1,85 milliard d’euros en crédits de paiement.

Nous soutenons évidemment ces dispositifs, qui contribueront très concrètement au renforcement de la continuité territoriale et au développement de l’emploi. Je tiens d’ailleurs à saluer l’effort global consacré à la continuité territoriale, qui voit ses crédits augmenter de plus de 41 %. C’est un message fort envoyé à nos concitoyens ultramarins, qu’ils soient étudiants ou actifs.

et la forte inflation qui y règne actuellement. Les efforts de ce budget 2024 portent essentiellement sur le logement – l’habitat insalubre reste bien sûr une priorité, tant le

les habitants de Mayotte sont contraints de recourir à des bouteilles d’eau en plastique pour leurs usages du quotidien, en l’absence de réhabilitation et d’accord local pour l’implantation d’un réseau rénové et sans fuite

et leurs nombreux rapports, ont permis cette évolution de crédits en faveur des Ultramarins l’Agence de l’outre mer pour la mobilité. Les crédits affectés au service militaire adapté progressent également chaque année. Ce dispositif d’insertion professionnelle de nos jeunes en décrochage scolaire est une belle réussite : à preuve, ses taux d’intégration à un emploi durable restent élevés.

Au titre de la politique de santé, les engagements de l’État demeurent inchangés, alors que le renouvellement de notre convention solidarité santé est toujours en attente. une promesse m’avait pourtant été faite l’an dernier dans cet hémicycle par votre prédécesseur, M. Carenco. Notre protection sociale est en difficulté

Au titre des aides à la reconversion de l’économie polynésienne, on note une stabilité des moyens délégués, dont les dépenses retenues portent sur le désenclavement des îles et sur la prévention des risques.

Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) voit ses crédits augmenter chaque année pour faire face au traitement des dossiers, de plus en plus nombreux, déposés par les victimes ou par leurs ayants droit. Il est très rassurant de voir l’État assumer ces réparations à un rythme soutenu depuis la mise en place du « 1 millisievert » – les chiffres le prouvent. Je tiens

ou encore, à La Réunion, de la crise des « gilets jaunes », qui y fut particulièrement rude, car nourrie par un profond sentiment d’exclusion des populations les plus précaires. À chacun des nombreux mouvements sociaux qui touchent les territoires d’outre mer, on retrouve les mêmes revendications

notre pays. Répondre rapidement et efficacement aux difficultés de pouvoir d’achat que rencontrent nos compatriotes d’outre mer est bien sûr un enjeu de cohésion sociale.

ont pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. Les OPMR donnent notamment un avis consultatif préalable à la phase de négociation des prix des produits composant le bouclier qualité prix. Mais ils sont contraints par le faible niveau de leur dotation, qui est d’environ 100 000 euros par an, et par la grande variété de leurs missions. Monsieur le ministre, dans l’intérêt du pouvoir d’achat de nos compatriotes d’outre mer, je vous propose d’augmenter significativement la dotation des OPMR.

seuls à même d’enclencher une dynamique vertueuse pour les outre mer. Monsieur le ministre, il faut travailler au développement d’une économie plus dynamique et durable, véritablement ancrée dans les territoires et plus respectueuse de son environnement, permettant une hausse du pouvoir d’achat des Ultramarins.

importateurs et distributeurs ; la taille des marchés locaux ; la fiscalité locale assise sur les importations ; le manque d’emplois locaux et la faiblesse des revenus ; ou encore l’insuffisance des productions locales, y compris pour les produits frais.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite ouvrir mon propos en paraphrasant notre Président de la République : les aéroports sont les lieux où se croisent les gens qui sont tout et ceux qui ne sont rien. Ceux qui sont tout bénéficient, entre autres, du privilège d’être nés au bon endroit. Ceux qui ne sont rien, nés à des milliers de kilomètres du continent, sont condamnés au chômage, à la vie chère, à la précarité, à l’eau boueuse et à l’exil. Réussir pour soi, chez soi, est de plus en plus difficile pour nous, chez nous, au nom du fallacieux argument de la rupture d’égalité, que l’on nous ressort à chaque fois

Malgré l’annonce de sa suppression, nous nous retrouvons aujourd’hui au Sénat pour continuer d’en débattre. N’avons nous donc rien appris de notre histoire ? Votre politique doit elle constamment être celle du grand bond en arrière ? Alors que l’outre mer souffre d’un taux de chômage qui est toujours au moins deux fois plus élevé qu’en Hexagone, vous avez eu l’idée – quelle révélation, quelle révolution ! – d’envoyer des travailleurs hexagonaux abonder nos entreprises et nos services publics.

S’il y a un dossier de mobilité à propos duquel nous avions des attentes, c’est bien celui de la continuité territoriale. Las ! une nouvelle fois, l’enveloppe allouée à l’ensemble des territoires ultramarins reste bien en deçà desdites attentes

Pourtant, avec nos 93 millions d’euros, nous faisons bien pâle figure à côté de la dotation annuelle de 187 millions d’euros allouée à l’île de Beauté.

nous pourrons toujours vous répondre qu’à Mayotte, où vous assurez la gestion partagée de cette même compétence, votre responsabilité a été pointée du doigt par l’Union européenne dans la crise que traverse le département.

Comme le disait Thomas Sankara, « il faut choisir entre le champagne pour quelques uns et l’eau potable pour tous ». Or le Gouvernement a fait son choix : le choix d’accepter qu’en France, pays des droits de l’homme, 2,7 millions de personnes, habitant trop loin du continent, soient susceptibles de manquer d’eau potable.

qui fait partie intégrante de la réalisation de tous les droits de l’homme ». L’outre mer représente 80 % de la biodiversité française. L’outre mer est notre puissance maritime. L’outre mer est la porte d’entrée de la France vers l’espace. L’outre mer est un berceau du multiculturalisme et de la laïcité. L’outre mer est un incubateur de nouveaux talents et d’innovation. L’outre mer porte en partie la jeunesse et le renouveau du pays. Mais l’outre mer, ce sont aussi des hôpitaux laissés à l’abandon ; des populations empoisonnées par la pollution des sols et des nappes phréatiques ; des descendants d’esclavagistes s’octroyant le privilège et les bénéfices d’un monopole sur nos économies. Dans les débats qui vont suivre, nous verrons que l’outre mer, c’est aussi la France des inégalités. La Réunion souffre d’une fracture sociale qui se répercute dans tous les pans de notre vie… faut conclure. Sans solution nouvelle pour le logement, sans contrôle ni des prix, ni des monopoles, ni des marges, ce sont des centaines de milliers d’Ultramarins que vous abandonnez à la misère ! Je vous prie de conclure. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre les crédits de cette mission.

France. Les problèmes de logement y amplifient de surcroît le déclin démographique, limitant d’autant les ressources disponibles pour assurer l’avenir de l’archipel et son adaptation au changement climatique. Pour 2024, le document de politique transversale relatif au budget de l’archipel affiche une augmentation de 1,522

réjouis. Bien sûr, ces rapports sont parfois tumultueux, mais je sais que nous parviendrons à avancer sur les chantiers qui nous attendent, dans l’intérêt de nos populations. Je salue évidemment

Comme vous le savez, indépendamment du contexte économique actuel, le problème du coût de la vie est structurel et persistant dans nos pays. C’est pourquoi je m’étonne de constater que, derrière la hausse globale des

débat d’amendements, de renforcer l’aide au fret en la complétant d’un nouveau volet fléché en direction des produits de première nécessité. Ainsi garantirait on à nos concitoyens des coûts accessibles, à l’heure où les écarts s’accentuent avec l’Hexagone, tirés en premier lieu par les prix de l’alimentation.

aidants. Le deuxième enjeu majeur de cette mission, c’est bien sûr le déploiement des nouveaux dispositifs relatifs à la continuité territoriale – vous m’en voyez ravie.

crédits est de soutenir les mobilités de nos concitoyens, qui sont parfois tenus éloignés de leur territoire et de leurs attaches du seul fait de leur condition sociale. Il y a là une violence

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, gouverner c’est choisir ses combats et c’est établir ses priorités. La mission « Outre mer » bénéficie, au sein du projet de loi de finances pour 2024, d’une hausse de ses crédits, dont je me félicite.

retard doit demeurer une priorité pour la France. Mais, nous le savons, tout ne peut pas se faire en un an. Le territoire de Saint Martin, que j’ai l’honneur de représenter à la Haute Assemblée, a besoin de cette solidarité nationale.

À cela s’ajoutent des handicaps structurels : une immigration importante, un chômage de masse – plus de 30 % –, une pauvreté endémique. Notre PIB par habitant, qui équivaut à 45 % du PIB par habitant hexagonal, fait de Saint Martin la troisième collectivité la plus pauvre de France ! Ces réalités sont peu connues, faute de statistiques

j’en suis convaincue, de refonder les cadres d’action de la politique du logement à Saint Martin, avec l’aide de l’État, par le biais de conventionnements sur des programmes spécifiques. C’est pourquoi je suis plus que favorable à l’adoption de l’article 55 de ce projet de loi de finances, qui permettra l’extension du périmètre d’intervention d’Action Logement à Saint Martin, conformément aux dispositions de la convention quinquennale 2023 2027 signée

Le problème du logement insalubre à Saint Martin justifierait cet effort supplémentaire, les besoins étant évalués par la collectivité à 2,5 millions d’euros par an. Plus de 5 400 résidences principales n’y sont pas raccordées au réseau de tout à l’égout, et seulement 39 % des ménages saint martinois disposent de l’eau chaude. En outre, afin de garantir un accès à l’eau potable et un traitement des eaux usées dans les normes pour tous les usagers ultramarins, il a été annoncé une révision et un renforcement du plan Eau DOM d’ici à six mois. Cette nouvelle mouture doit intégrer les nouvelles mesures du plan Eau annoncées par le Président de la République le 30 mars dernier,

Saint Martin continue de s’inscrire dans une logique de rattrapage et l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint Martin (EEASM) reste dépendant des subventions publiques pour le financement de ses investissements, lesquels devront être amplifiés durant la prochaine décennie. décennie. Certes, dans un contexte très difficile, l’EEASM est parvenue à investir en moyenne 9,3 millions d’euros par an au cours de la période 2016 2020, mais cet effort devra être renforcé : dans les dix prochaines années, il faudra à tout

Merci